Je pense notamment à une famille de ma commune qui m'a contactée ce week-end : elle souhaiterait reporter un mariage, initialement prévu le 18 juillet prochain, mais le prestataire leur a indiqué qu'une demande de report serait considérée comme une annulation et qu'il n'y aurait pas de remboursement d'acompte.

prestataire ? D'autres questions se posent : les réunions de personnes qui peuvent être limitées ou interdites par décret seront-elles autorisées ? Les citoyens venant d'autres départements ou d'autres pays pourront-ils se déplacer pour assister à un mariage ?

Encore faut-il que ces mesures soient effectivement exceptionnelles et, bien sûr, temporaires. Encore faut-il être sûr qu'elles disparaissent avec l'état d'urgence lui-même. Nul n'a oublié ces dispositions de l'état d'urgence de 2015 entrées finalement dans le droit commun. L'état d'urgence est un outil, ne nous y installons pas. Il ne pallie pas les manquements que la pandémie a rendus plus criants encore, à commencer par ces choix austéritaires et libéraux successifs en matière de santé publique qui ont mis nos hôpitaux dans l'état où ils sont aujourd'hui. Le confinement a été mis en place d'abord pour éviter leur possible engorgement. Ce sont aussi les choix économiques de nos dirigeants qui ont fragilisé notre industrie. Nous sommes dépendants notamment de la Chine pour ces masques, qui n'arrivent pas, pour ces tests, qui ne sont pas prêts, pour ces respirateurs, qui ne sont pas aux normes ; sans compter le manque de médicaments et de blouses pour nos soignants. Cette pandémie a été affrontée dans la confusion, avec des contradictions multiples et pas mal d'amateurisme. Le déconfinement semble prendre le même chemin. Nous voulons plus de masques, plus de tests, plus de lits. L'état d'urgence n'est pas la priorité, il sert juste de bouclier à l'exécutif.

Il vise à préparer dès aujourd'hui une sortie dégressive de l'état d'urgence sanitaire sans repousser le débat au 10 juillet, ce que nous saluons. Depuis l'expérience de l'état d'urgence déclenché après les attentats de 2015, nous savons à quel point il est difficile de sortir de ces régimes dérogatoires du droit commun. Il se produit une sorte d'effet cliquet d'accoutumance aux latitudes permises par ces régimes. Afin de ne pas reproduire cette expérience et de faire émerger plus rapidement la question de l'adaptation structurelle du droit existant, notre collègue propose un dispositif en deux temps dans un premier temps, l'état d'urgence sanitaire serait maintenu de façon intégrale ; dans un second temps, le Gouvernement pourrait seulement avoir recours aux mesures prévues aux 3°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les plus opérationnels du point de vue de la gestion de crise. De façon générale, cet amendement invite à repenser les régimes d'urgence pour l'avenir, dès lors que des sas de sortie pourraient être aménagés dès leur conception législative. C'est la raison pour laquelle je le défends aujourd'hui. Il vise ainsi à retrouver plus rapidement un exercice normal des libertés auxquelles le groupe du RDSE est par tradition très attaché. En outre, il tient compte de la facilité avec laquelle l'état d'urgence sanitaire pourrait être établi en cas de seconde vague, tel que le prévoit le régime adopté le 23 mars dernier. L'amendement

Rappelons que, si nous sommes confinés depuis bientôt deux mois, c'est en raison de l'impréparation du Gouvernement et de son incapacité à gérer dans l'urgence notre approvisionnement en masques de protection et la mise en place d'un dispositif de dépistage qui aurait permis de ne pas ajouter au chaos sanitaire un chaos économique et social. C'est l'anticipation qui a manqué hier pour sauver des vies. C'est le temps qui manque aujourd'hui pour faire parvenir à chacun le nécessaire pour reprendre une activité professionnelle normale. On gagne du temps quand on prévoit. On gagne du temps quand on gouverne. Mais quand le temps est perdu, il ne se rattrape jamais. Le temps, c'est des vies sauvées ou des vies perdues. Les hésitations, les mauvaises décisions et, trop souvent, les mensonges nous ont fait perdre beaucoup de temps et donc beaucoup de vies. Aujourd'hui, il nous semble disproportionné de proroger pour deux mois, sans visibilité. Je propose de proroger d'un mois et de revenir, le cas échéant, sur le terme prévu. L'urgence est de rendre à la société et à nos compatriotes leurs libertés publiques et aux entreprises leur travail dès le mois de juin, à condition, bien de s'en donner les moyens. Les dispositions de cet amendement prévoient également un contrôle du Parlement d'ici à un mois pour juger des suites à donner à cet état d'urgence. En effet, si le Gouvernement profite de l'actualité pour amnistier ses proches ou enterrer la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla,

Pourquoi ? Parce que nous travaillons dans des conditions exorbitantes jamais vues. Parce que, depuis un mois, voire davantage, les injonctions du Gouvernement sont tellement contradictoires, tellement changeantes, la situation tellement variable

date au 10 juillet, souhaitant ainsi pouvoir se prononcer, si besoin était, dans un délai plus court que celui proposé par le Gouvernement. Cette demande tout à fait légitime semble satisfaite par les dispositions de notre amendement, qui tend à inclure dans la période d'état d'urgence sanitaire le week-end précédent et le jour de la fête nationale, ce qui permet de faire correspondre l'état d'urgence sanitaire avec l'échéance de la mi-juillet évoquée par le Président de la République. La levée de l'état d'urgence sanitaire juste avant le 14 juillet pourrait laisser penser que les restrictions imposées d'ici là seraient abandonnées, ce qui entraîne une incertitude prolongée et une imprévisibilité pour les Français, notamment pour les élus locaux organisateurs des festivités durant ce week-end.

des acteurs publics et privés en cas d'infraction non intentionnelle. Vous connaissez bien ce dispositif, puisqu'il s'agit de la loi Fauchon : lorsque le lien de causalité avec le dommage est indirect, la responsabilité pénale ne peut être engagée

que les décideurs publics seraient irresponsables. En deuxième lieu, la commission entend modifier le régime de la responsabilité pénale pour les seuls faits

la commission, tel qu'il est formulé, donne l'impression que le premier pourra être poursuivi pour imprudence ou négligence, alors que le second ne pourra l'être qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une mesure

Mais comment ne pas entendre ce que nous disent les élus locaux tous les jours ? Ils n'ont pas été associés à la définition des règles relatives à l'ouverture des écoles,

Gremillet, que la responsabilité pénale du maire et des directeurs d'école ne puisse pas être engagée dans trois situations : lorsqu'ils sont amenés à évaluer dans un temps très court la capacité d'accueil des élèves dans un établissement scolaire

Ce matin, nous avons fait deux choses. D'abord, nous avons considéré que, si le Gouvernement voulait reconduire une nouvelle fois l'état d'urgence, il faudrait qu'il revienne devant le Parlement avant le 23 juillet

: nous ne pouvons jamais écarter la mise en cause de la responsabilité pénale d'une personne qui aurait intentionnellement provoqué une contamination, ni admettre qu'on exonère de sa responsabilité pénale une personne qui aurait commis, par violation délibérée d'une obligation particulière de prudence imposée par les lois et les règlements, un acte ayant entraîné une contamination.

pour le motif qu'elle aurait commis une faute caractérisée parfaitement indéfinie dans le code pénal, mais que le juge invoquerait pour rechercher la responsabilité pénale de cette personne qui, du fait de la politique du Gouvernement, aurait pris un risque.

: inspiré par de nombreuses remarques des maires du département de l'Eure, qu'il a à coeur de défendre, il a pris très tôt des initiatives pour faire avancer la réflexion.

combien d'autres dispositions ne devrions-nous pas aussi introduire dans la loi ? Il y a un moment où c'est trop ... D'autant qu'on nous reproche, à juste titre, de faire des lois trop bavardes. Laissons à chaque échelon de responsabilité ses propres attributions.

de loi. Vous écrivez dans l'objet de cet amendement qu'il serait difficile de mesurer dans l'urgence les conséquences d'une telle restriction de la responsabilité pénale. Mettez-vous donc un peu à notre place Nous avons découvert samedi après-midi un projet de loi dont je ne veux pas exagérer l'importance, mais qui, tout de même, comporte des dispositions mettant en cause le respect de la vie privée, le secret médical et un certain nombre d'autres garanties et libertés. Or vous ne nous avez pas entendus dire qu'il nous était difficile de nous prononcer, parce que nous faisons notre devoir. Nous préférons, bien sûr, avoir du temps, comme vous préférez en avoir. Ne disqualifiez donc pas notre travail au motif que vous n'auriez pas eu le temps de réfléchir, alors que l'exécutif, jusqu'au plus haut niveau de l'État,

Nous limitons, dites-vous, cette disposition pénale aux faits commis pendant l'état d'urgence sanitaire. Mais, madame la garde des sceaux, nous l'avons fait exprès ! C'est justement parce qu'il y a l'état d'urgence sanitaire, une situation exceptionnelle, qu'il nous faut, pour la traiter,

différentes ! Et si l'état d'urgence sanitaire n'est pas une situation différente justifiant l'application d'un droit différent- à condition

de le retirer. Nous pourrons ainsi poursuivre le travail que nous avons commencé sur les bases que nous avons définies, des bases dont j'ai la faiblesse de croire qu'elles ont été précédées d'une réflexion approfondie et qu'elles ont abouti à un résultat équilibré.

de la disposition que nous prenons sur la responsabilité pénale, notamment des maires, il faut dire à nos élus, pour les rassurer, qu'ils n'ont, d'après la loi, aucune décision à prendre pour l'ouverture des écoles, car l'article L. 411-1 du code de l'éducation nationale prévoit que cette responsabilité incombe aux directeurs et directrices d'école, sous l'autorité des inspectrices et inspecteurs d'académie. Le maire, bien sûr, fait partie du conseil d'école et fournit des moyens. Si ces moyens n'étaient pas suffisants pour assurer la sécurité sanitaire

pour vous expliquer les raisons pour lesquelles nous sollicitons la prolongation de cet état d'urgence assez extraordinaire, caractérisé par une restriction des libertés liée à la volonté de protéger la santé des Français. J'y insiste, nous appuyons nos décisions sur l'avis des scientifiques.

alentours du 10 mars. Cependant, il s'est passé depuis des choses extrêmement éprouvantes, avec plus de 20 000 morts dans notre pays, des hôpitaux encore très chargés, qui ont frôlé la sursaturation, mais qui ont tenu et qui ont besoin d'un peu plus de temps.

Madame la garde des sceaux,

Je sais bien qu'il n'y a pas de rupture d'égalité quand on traite différemment des situations différentes, mais je veux dire ici que nous ne sommes pas nécessairement dans une situation différente au regard du Covid-19,

qu'il est très important de prendre en compte la nécessité des circonstances spécifiques liées à la crise sanitaire. Il est possible de le faire, mais dans un dispositif global, valable pour l'ensemble des décideurs publics

alors même que leur légitimité démocratique est fragilisée par la non-installation, au nom de la crise sanitaire, des conseils

protocole sanitaire apocryphe arrivé par des voies assez surprenantes et dont on leur a dit, quelques jours plus tard, qu'il n'avait aucune valeur. Ce week-end, ils ont dû digérer un autre protocole, mesurer la différence

que ces moyens puissent exister dans les écoles maternelles et élémentaires. Ils n'ont jamais existé. Nettoyer, tous les jours, les stylos utilisés par les enfants répond à un protocole totalement hors sol,

! Entre le protocole apocryphe où le repas devait être distribué dans les classes et le protocole authentifié, on a changé dix fois de mode d'organisation. Or la responsabilité des maires est engagée, ... Il faut

à notre très estimé président de la commission des lois ... Premièrement, il n'est absolument pas question de placer les élus au-dessus de la loi. Il n'est absolument pas question de préparer

commission, qui est désormais intégré dans le texte, tout simplement parce que nous sommes sur une matière qui est évolutive. Vous savez, parce que vous êtes juriste,

D'abord, personne ici, pas plus à droite qu'à gauche, n'a le monopole du coeur à l'égard des élus. Nous sommes tous conscients de l'inquiétude de ces derniers. Elle remonte de chacun de nos départements,

C'est la raison pour laquelle, à mon grand regret, mais aussi en cohérence avec la tribune que nous avons signée hier et la position que nous avons défendue dans les questions qui vous ont été posées aussi bien aujourd'hui que les jours précédents, le groupe La République En Marche ne votera pas l'amendement du Gouvernement.

et, surtout, adapter leurs services municipaux pour appliquer les décisions de l'État dont ils sont les délégataires. Aujourd'hui, il convient non seulement de reconnaître l'importance de leur investissement d'élus dans l'application de la directive du ministère, mais aussi, et surtout, de reconnaître leur responsabilité morale. Qu'adviendra-t-il de l'esprit d'un maire si un cas de contagion était reconnu dans l'école communale dont il a la charge ?

: « Juste une remarque sur la responsabilité des maires. Pour ma part, je prépare la réouverture de mon école. J'ai les masques. Nous travaillons avec l'école sur l'organisation à mettre en place. Quelques maires se préparaient aussi à cette réouverture. Mais la lecture ce week-end du protocole sanitaire les interroge davantage quant à leur responsabilité. Certains sont prêts à faire machine arrière s'ils n'ont pas de réponse

recourir au télétravail si c'est possible et fournir des masques et des gels. Face à ces obligations, l'employeur court des risques d'être assigné devant le conseil des prud'hommes pour manquement à la sécurité. Actuellement, le code du travail ne prévoit pas d'obligation particulière liée à l'épidémie de Covid-19. En revanche, les dispositions du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoient qu'afin de ralentir la propagation du virus « les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites " barrières ", définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance Indiscutablement, ce décret est un règlement au sens précité et impose à tout un chacun, salariés comme employeurs, une obligation qui consiste à respecter des gestes barrières. Toutefois, il ne définit pas les mesures d'hygiène, ni le principe de distanciation sociale. Ainsi, la formulation des dispositions relatives à la mise en danger d'autrui, les prévisions du décret ne sont à l'évidence pas suffisamment précises pour permettre à l'employeur de connaître les mesures qu'il doit mettre en oeuvre pour protéger les salariés et, partant, partant, de savoir à quel moment il s'écarte de façon « manifestement délibérée » de ses obligations et met volontairement ses salariés dans une situation de danger. Cela étant, les salariés aussi ont une obligation quasi juridique : protéger leur santé et celle d'autrui. La non-pratique des gestes barrières, se laver les mains, prendre du gel hydroalcoolique et porter un masque quand c'est obligatoire, peut entraîner des plaintes à leur encontre venant de l'employeur ou d'autrui qui peut en être victime.

Nous considérons que, dans ce cadre, nous obtenons beaucoup d'explications du Gouvernement, soit oralement lors des auditions, soit en écrivant aux ministres, qui répondent en général très rapidement ; d'ailleurs, nous ne manquons pas de les relancer quand ce n'est pas le cas. le Premier ministre a répondu à la commission des lois sur son premier rapport d'étape. Je lui ai de nouveau écrit la semaine dernière, et il ne manquera pas, j'en suis certain, de me répondre.

est à M. Jérôme Durain. La gestion de la crise sanitaire dans les territoires est une affaire de couple. On nous a beaucoup présenté le couple maire-préfet comme le garant des bonnes conditions du déconfinement. Mais il est un autre couple qui compte : le couple président du conseil départemental-préfet. Nous sommes tous conviés à des réunions, souvent informelles, qui se tiennent selon des configurations variées, avec les parlementaires, le préfet, les maires, les représentants des associations d'élus. Pourtant, rien ne vient formaliser cette coopération. cette coopération. Cela fait peser sur les maires une responsabilité qui peut dépasser leurs compétences et qui ne correspond pas à la part qu'ils ont prise dans les décisions venant de l'État. conséquent, cet amendement vise à mettre en place un protocole particulier entre le maire et le préfet, ce qui est une demande de l'Association des maires de France. Pour clarifier, encadrer et rendre plus efficace la coopération que j'évoquais, nous ajoutons un protocole particulier entre le préfet et le président du conseil départemental. Enfin, nous souhaitons que les groupements de communes, dont le rôle est essentiel dans la gestion de la crise sanitaire, soient associés à ces deux protocoles particuliers.

de reprise des cours. Nous avons eu un débat très intéressant et parfaitement légitime sur la responsabilité des élus locaux, en particulier des maires, et sur la nécessité de les sécuriser

la conformité au protocole prescrit par le ministère de l'éducation nationale des conditions d'accueil et des mesures sanitaires mises en place dans chaque école. La responsabilité qui incombe au maire

par les parents puisse être évoquée avec l'ensemble de la communauté éducative. Enfin, le transport scolaire, indispensable à la réouverture des classes, devant être sécurisé, il est également proposé qu'un règlement y afférent soit validé par les représentants du ministère de la santé et de celui des transports.

Dans la continuité des lois et ordonnances précédentes qui ont rogné le droit du travail, l'état d'urgence sanitaire a servi d'excuse au Gouvernement pour affaiblir encore davantage les protections collectives, en remettant en cause les durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos. Ces règles protectrices sont des acquis importants, essentiels pour la santé et la sécurité des salariés.

L'objectif sanitaire, que nous sommes censés partager, est la protection de l'ensemble de la population, en particulier des salariés qui ont repris ou vont reprendre leur activité professionnelle. Dérégler les temps de travail et faire exploser le seuil des 40 heures expose la santé des salariés à des conséquences extrêmement négatives, comme en attestent toutes les études.

Nous avions alerté sur les dangers des dispositions adoptées lors de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, et nous ne nous étions malheureusement pas trompés. Telle est la réalité des conditions de travail et des relations dans les entreprises

de cet amendement, nous tentons une nouvelle fois de rétablir les prérogatives du Parlement dans cette période d'état d'urgence sanitaire. Actuellement, la possibilité pour le Parlement d'interrompre par un vote l'état d'urgence sanitaire n'est pas prévue.

Rappelons que les catégories d'état d'urgence déjà appliquées de 1955 à 2015 prévoyaient que toute prorogation devait s'accompagner de la détermination d'une date de fin de l'état de crise.

pour éviter tout abus de pouvoir d'un exécutif s'appuyant sur une majorité qui ne prendrait pas en compte cet élément essentiel pour la démocratie,

ou de résolution ou un débat relatif à l'état d'urgence soit inscrit par priorité à l'ordre du jour, sur l'initiative de la conférence des présidents de chaque assemblée, pendant la session

articles 16 et 36 de la Constitution. Je ne comprends donc ni votre réticence aujourd'hui à permettre une telle intervention du Parlement ni votre acceptation de la mise en oeuvre de cet état d'urgence d'exception dépourvu de date butoir. Nous insistons, une fois encore, sur l'impérieuse nécessité de limiter clairement la durée de l'état d'urgence, sanitaire ou pas. Nous vous proposons d'armer le Parlement pour imposer la cessation d'une forme de pleins pouvoirs, dangereuse pour la démocratie. Quel

pour une durée d'un an, pendant laquelle le Gouvernement pourra décider d'interrompre la mise en oeuvre des mesures de l'état d'urgence ou de les reprendre par décret, ce qui devra alors donner lieu, au bout d'un mois, à un vote

Robert Laufoaulu, je souhaite appeler attention du Gouvernement sur la situation spécifique de Wallis-et-Futuna, où la sortie du confinement suscite de grandes inquiétudes. Ce territoire était, grâce à la fermeture des liaisons extérieures, épargné par la pandémie, fort heureusement car le système sanitaire et hospitalier y est peu développé et de nombreux habitants souffrent déjà de lourds problèmes de santé, comme le diabète.

Pourriez-vous cependant, monsieur le ministre, rassurer les populations de Wallis-et-Futuna et nous donner des précisions sur la volonté de l'exécutif d'apporter toutes garanties pour protéger les habitants et faire

Cette déclaration est surprenante à deux titres. D'une part, le virus circule énormément dans un certain nombre de pays de l'espace Schengen. À quel titre les ressortissants de ces pays se verraient-ils

une nouvelle fois en appeler à l'esprit de responsabilité. Aujourd'hui, le Gouvernement demande aux entreprises de poursuivre le télétravail et d'adapter les horaires des salariés devant se déplacer, afin de limiter l'encombrement des réseaux. Pour autant, ce n'est rien de plus et rien de moins qu'un simple appel à la bonne volonté et à l'esprit civique, sans incitation ni sanction. De l'autre côté, les usagers des transports sont soumis à de réelles obligations, notamment celle de porter un masque durant leurs trajets. Par ailleurs, les entreprises et les autorités organisatrices devront faire respecter aux usagers des règles permettant de garantir la distanciation sociale et les gestes barrières, en limitant les possibilités d'occupation des véhicules,

comment se satisfaire d'une obligation de port de masque qui ne serait pas adossée à un réel droit au masque gratuit, pour les usagers comme pour le personnel ? Comment se contenter d'un appel à la bonne volonté des entreprises pour limiter l'engorgement des transports collectifs, dans les régions les plus denses, notamment l'Île-de-France ?

seul maître à bord ; aucune disposition concrète n'est prévue pour limiter effectivement la demande de mobilité. Il s'agit pourtant d'une condition incontournable pour permettre le respect des gestes barrières. Comment garantir la sécurité du personnel dans ces conditions ? Quels droits pouvons-nous donner aux salariés quand les wagons, à n'en pas douter, vont rester trop fréquentés pour limiter la propagation du virus ? Ce flou entretenu témoigne d'une difficulté à faire réellement primer les enjeux de santé sur les enjeux économiques de reprise de l'activité « quoi qu'il en coûte

nous conduire à remettre en cause le dogme de la concurrence libre dans les transports urbains. On voit bien que la multiplication des acteurs rend plus difficile et complexe la réaction en temps de crise. Autant de pistes de travail, mes chers collègues, que nous

En Île-de-France, les transports en commun, empruntés avant la crise sanitaire par 5 millions de voyageurs chaque jour, sont susceptibles de constituer un goulet d'étranglement lors du déconfinement. Afin de ne pas saturer le système de transport, ce qui contribuerait à relancer une nouvelle vague épidémique, il est nécessaire de limiter les déplacements au moyen de la mise en place d'une attestation de déplacement dont le principe serait calqué sur l'attestation de déplacement dérogatoire aujourd'hui en vigueur en période de confinement. d'insérer dans le texte pourra notamment préciser que les attestations délivrées par les employeurs viseront à lisser les déplacements sur plusieurs plages horaires.

Pour tous les pratiquants, quelle que soit leur religion, cette pratique n'est pas accessoire, mais essentielle, au sens étymologique du terme. La liberté religieuse ne peut être assimilée à un loisir superflu.

monsieur le président.

a accepté de faire évoluer sa position, qui renvoyait à l'origine la réouverture des lieux de culte au mois de juin : il nous a indiqué que la date du 28 mai était désormais à l'étude. On se rapproche donc

à un dialogue approfondi avec les représentants des cultes. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de leur demander d'être auditionnés par la commission des lois.

pas d'autorité, mais venant en quelque sorte consolider les propositions d'organisation que chaque culte serait amené à faire de manière que le déroulement des cérémonies soit tout à fait compatible avec les exigences de sécurité sanitaire.

Or ce cimetière était pour lui un lieu symbolique : il y allait chaque jour mener un dialogue très singulier, au-delà de la mort, en se recueillant sur la tombe de son épouse.

de produire. Les pratiquants, quelle que soit leur religion, ne sont pas des citoyens de seconde zone ; entrer dans une église, une synagogue ou une mosquée

le confinement, beaucoup d'artistes ont joué et jouent encore un rôle précieux auprès de nos concitoyens, en leur permettant de s'évader par la pensée.

L'intermittence ne couvre en effet qu'une partie des contrats de toutes les professions du secteur culturel. Ainsi, pour l'ensemble du secteur, la réouverture paraît être l'aide la plus efficace.

actuelle du code de la santé publique autorise la réquisition, par décret réglementaire, de toute personne nécessaire au fonctionnement des services et à l'usage des biens nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire.

Guillotin. Le présent amendement vise à préciser davantage le cadre des réquisitions de personnes destinées à former les brigades médicales. Il paraît en effet nécessaire de prévoir dans la loi que ces personnes qui auront à collecter des données médicales sensibles soient bien qualifiées pour le faire.

jour. Il recommande la réquisition de services de restauration pour trouver des solutions d'aide alimentaire à destination de ces enfants. Cet amendement vise donc à permettre aux maires de solliciter le préfet pour envisager de telles réquisitions. Quel

brigades sanitaires », expression inspirée d'une formule du professeur Delfraissy, reprise par le Gouvernement pour expliquer qu'on allait mobiliser un certain nombre d'agents afin de remonter

Je ne vois pas vraiment de raisons de restreindre à ces brigades sanitaires, qui n'ont pas de statut particulier, la réquisition

de vote. Jérôme Durain a très bien fait de soulever ce problème de méthode politique et de comportement,

sociale. L'état d'urgence sanitaire ne peut avoir pour conséquence d'affamer les plus vulnérables de notre société. Assurer que nos concitoyens qu'ils ne souffriront pas de la faim durant l'épidémie doit faire partie de l'arsenal des mesures visant à garantir la santé publique pendant l'état d'urgence sanitaire.

recrudescence des besoins en matière d'aide alimentaire démontre que l'état d'urgence sanitaire est aussi un état d'urgence sociale ; le Gouvernement se doit d'y répondre.

négatif n'est pas une garantie absolue que la personne n'est pas porteuse du virus et qu'elle ne va pas contaminer d'autres individus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous allons demander à tous nos concitoyens

Depuis un mois, une opération de mise à l'abri de la population migrante a été déployée dans le Pas-de-Calais, mais cette mesure repose sur le volontariat, ce qui ne permet pas d'atteindre les objectifs sanitaires visés.

que les résidents de Corse. Nous pensons notamment aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont contraints de transiter par le Canada pour rejoindre la métropole faute d'offre de transport aérien direct. Introduire une différence entre les territoires d'outre-mer, souvent insulaires, nous paraît totalement injustifié. L'amendement

vise à étendre les mesures de confinement aux personnes en situation irrégulière déjà présentes sur le territoire national. Cette disposition trouverait une application toute particulière dans les territoires touchés par la crise sanitaire et connaissant un afflux important de personnes en situation irrégulière, dont la mise à l'abri sur la base du volontariat n'a pas été efficace. Ainsi, dans les Hauts-de-France, le Calaisis connaît un regain de tensions dû à la pression migratoire dans un contexte de crise sanitaire. Les déplacements de personnes en situation irrégulière qui ne peuvent pas respecter les consignes sanitaires- mesures de distanciation sociale et gestes barrières -laissent craindre une propagation plus rapide de l'épidémie, malgré le respect des mesures par l'ensemble Il semble indispensable que l'État prenne ses responsabilités afin de faire respecter les consignes sanitaires à des populations démunies et de rassurer les habitants du Calaisis. L'amendement

pour protéger la population contre les risques de contamination. C'est la raison pour laquelle je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.

La réussite de la levée du confinement est conditionnée, entre autres choses, au respect scrupuleux et potentiellement contraignant, par les personnes atteintes et les personnes contacts, d'un isolement prophylactique à domicile ou à l'hôtel, selon le risque de reconstitution de foyer. Limiter l'isolement prophylactique à une simple recommandation médicale dénuée de tout effet contraignant ne prémunit absolument pas le pays contre le surgissement d'une seconde vague épidémique, à laquelle notre système hospitalier ne manquerait pas de succomber. Mon amendement a pour objet d'étendre les cas dans lesquels le préfet se verra habilité, par décret du Premier ministre instrumentant l'état d'urgence sanitaire, à arrêter des mesures individuelles individuelles de mise en quarantaine et d'isolement, en ajoutant celui d'un refus réitéré d'une mesure médicale et individuelle d'isolement prophylactique.

monsieur le président de la commission des lois.

mais pour des personnes qui ne respecteraient pas les prescriptions qui leur auraient été faites

est attendu en raison du civisme de nos compatriotes, de leur esprit de responsabilité, de leur sens du devoir à l'égard d'autrui. Qu'est-ce

Personnellement, je ne les trouve pas excellents. Vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre, l'épidémie est toujours là. Actuellement, les services de réanimation ne sont plus en tension comme ils ont pu l'être, mais il suffirait de peu de choses pour qu'ils le redeviennent, avec bien sûr des disparités géographiques. On sait

Malgré des motifs réels d'hésitation, je défends la proposition du président Milon et je n'adhère pas à une partie du raisonnement présenté par Philippe Bas. Il n'y a pas d'opposition entre

à l'ordre nécessaire les personnes qui choisissent délibérément de s'opposer aux mesures d'isolement. L'argument du président Bas est de dire qu'il y aura des difficultés d'application. C'est indéniable, comme pour tous les systèmes de contrôle. Mais la démonstration qu'il a avancée est trop systématique.

se voit recommander, par un médecin ou par la plateforme de l'assurance maladie, de rester chez lui, ni la police ni la gendarmerie n'en sont évidemment informées.

Il n'empêche que l'immense majorité de la population française a respecté scrupuleusement le confinement, jusqu'à faire baisser le taux de transmission du virus à 0,5, soit le plus bas taux d'Europe. Encore une fois, toute notre stratégie repose sur la confiance, l'explication, la pédagogie, le soin, l'attention portée à l'autre.